Au cours de l'année passée, monsieur le Premier président, vous vous êtes personnellement rendu à plusieurs reprises devant nos commissions des finances et des affaires sociales pour présenter les travaux de la Cour, qui jalonnent la préparation et l'exécution des lois financières.

le recours aux contractuels dans l'éducation nationale, les équipements de la police et de la gendarmerie, les conditions de versement des aides agricoles ou, tout récemment, la prise en charge des victimes du terrorisme.

De manière plus générale, la Cour est régulièrement sollicitée par les commissions et délégations de notre assemblée, et je crois pouvoir dire- ce n'est pas simplement un propos de courtoisie -que ses travaux constituent un apport précieux dans l'exercice de notre fonction de contrôle comme de notre fonction législative.

Il intervient cette année dans un contexte encore incertain pour les finances publiques, comme nous avons pu le constater dans les derniers jours de la discussion budgétaire- nous l'évoquions ensemble avant cette séance solennelle. Cela renforce d'autant l'attention que nous devons porter aux observations de la Cour en matière de gestion des administrations et organismes publics. Monsieur le Premier président, nous allons à présent vous écouter présenter le rapport annuel de la Cour des comptes, puis nous entendrons le président de la commission des finances et le président de la commission des affaires sociales. Je vous laisse donc

monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, la parution de notre rapport public annuel est devenue, pour les juridictions financières, un rendez-vous phare avec les Français. En complément des travaux publiés tout au long de l'année, elle nous conduit à réaliser à leur intention un exercice d'explication et de pédagogie sur une grande variété de sujets, conformément à la mission d'information que nous a confiée le constituant, en leur fournissant des éléments objectifs, objectifs, étayés, contredits, vérifiés et s'appuyant sur des comparaisons internationales toujours utiles, même si elles ne sont pas systématiquement reproductibles. La publication de ce rapport annuel est aussi un temps fort, vous l'avez rappelé, monsieur le président, dans les relations déjà très denses que nous entretenons avec la représentation nationale. En plus de celui-ci, le Parlement est en effet destinataire d'un grand nombre de nos travaux tout au long de l'année. Certains viennent spécifiquement alimenter la procédure d'examen des textes financiers, en application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et de la loi organique relative aux lois de financement de de la sécurité sociale. Ils font ainsi pleinement vivre la mission d'assistance confiée par l'article 47-2 de la Constitution à la Cour des comptes, au bénéfice, notamment, du Parlement dans son activité de contrôle du Gouvernement. L'Assemblée nationale et le Sénat

concertée, la programmation de leurs travaux que les juridictions financières établissent en toute indépendance. Les rapports réalisés dans ce cadre portent sur des politiques publiques stratégiques, à forts enjeux. En 2018, la commission des finances de votre assemblée a reçu, par exemple, communication d'enquêtes portant sur le soutien aux énergies renouvelables, l'indemnisation des victimes du terrorisme ou les matériels d'équipement dans la police et la gendarmerie. En tout, ce sont ainsi douze enquêtes qui ont été réalisées à la demande des assemblées parlementaires. Elles s'ajoutent aux très nombreux travaux effectués par les juridictions financières qui vous sont transmis chaque année : rapports publics thématiques, notes d'exécution budgétaire, actes de certification, référés, rapport sur les finances locales ... Le total, pour pour 2018, s'élève à 190 travaux qui vous ont été adressés. Le troisième tome de notre rapport public annuel vous en donnera un détail plus complet. J'ajoute que, au cours de cette même année, la Cour a été auditionnée à 80 reprises par le Parlement. Je me réjouis évidemment de ces chiffres. Surtout, je souhaite que la quantité très importante d'informations qui vous est transmise de notre part soit aussi utile que possible à l'exercice de votre mandat. J'en viens à présent aux trois principaux messages que notre rapport public annuel formule. Le premier porte sur la situation de nos comptes publics. La Cour constate, d'une part, la fragilité du redressement opéré ces dernières années elle relève, d'autre part, les incertitudes qui pèsent sur la trajectoire des finances publiques pour les mois à venir. Dans un cadre budgétaire contraint par l'état de nos comptes, notre pays doit amplifier et systématiser la modernisation de ses services publics pour les rendre plus efficaces et plus efficients. En la matière, des possibilités existent ; elles sont même nombreuses. C'est le deuxième message de ce rapport. Il n'est en rien nouveau- je l'ai d'ailleurs formulé devant vous à de nombreuses reprises -, mais il est, je crois, essentiel de le réitérer dans le contexte que connaît notre pays et qui pousse, parfois, à la résignation. Pour redonner du souffle à nos comptes et pour alléger le poids de notre dette, notre rapport identifie, comme l'ont fait ses précédentes éditions, des marges d'économies et de ressources nouvelles. Certaines de ces marges sont déjà connues ; elles rejoignent d'ailleurs parfois des propositions que vous formulez dans vos travaux d'évaluation et de contrôle. Mais les actions tardent souvent à venir ou à porter pleinement leurs fruits. Aussi notre rapport esquisse-t-il, au travers d'exemples de transformations réussies comme, à l'inverse, de situations d'immobilisme, quelques conditions à remplir pour se saisir des opportunités de modernisation de l'action publique s'offrant aux décideurs. Ce sera mon dernier message. Je dirai quelques mots, à présent, sur chacun de ces messages. Chaque année, la parution du rapport public annuel est l'occasion de porter une appréciation sur l'état de nos finances publiques. S'agissant de 2018, la Cour constate d'abord que le redressement de nos comptes publics semble marquer le pas. Après huit années ininterrompues de baisse, le déficit public s'établirait à un niveau proche de celui de 2017, soit à 2,7 points de selon la dernière prévision fournie par le Gouvernement. Cette prévision semble réaliste, voire prudente, compte tenu des données actuellement disponibles. Elle ne pourra toutefois être confirmée que par les résultats complets de l'exécution budgétaire pour l'année 2018, qui, comme vous le savez, ne seront disponibles qu'à la fin du mois de mars. Nous aurons l'occasion d'approfondir ces premières analyses lors de la remise des rapports sur l'exécution du budget de l'État et sur la situation et les perspectives des finances publiques. Nous le ferons cette année en expérimentant un calendrier renouvelé, qui vous permettra de disposer avant l'été de l'ensemble des analyses des juridictions financières sur l'exécution budgétaire portant sur l'année passée, comptes sociaux

le solde structurel de nos comptes. Le déficit structurel pour 2018 devrait se maintenir au niveau atteint en 2017, soit autour de 2,3 points de PIB, selon le Gouvernement. Mécaniquement, cette situation devrait accroître notre dette publique, dont le montant approcherait 98,7 % du PIB. Derrière les chiffres, ce que je veux souligner devant vous, c'est le décalage qui continue de se creuser entre la France et la majorité de ses partenaires européens. La plupart d'entre eux font en effet beaucoup mieux. En moyenne, la dette publique des pays de la zone euro pour 2018 est ainsi inférieure, de plus de 10 points de PIB, à celle de la France. La dette publique allemande, pour sa part, n'a cessé de se réduire depuis 2012 et approche désormais le seuil de 60 du produit intérieur brut. Ce pays va ainsi quasiment revenir au niveau de dette qui était le sien- et qui était aussi le nôtre ! -en 2007. Dans ce premier chapitre, la Cour formule également une appréciation sur l'évolution des finances publiques nationales pour 2019. Cette dernière apparaît, à bien des égards, très incertaine. Permettez-moi un bref rappel des circonstances que vous connaissez. La trajectoire inscrite en septembre 2018 dans le projet de loi de finances qui vous a été présenté a été substantiellement modifiée par les mesures d'urgence annoncées en décembre, en réponse au mouvement des « gilets jaunes Le projet de loi de finances initiale pour 2019 anticipait une dégradation du déficit public, le fixant à 2,8 points de PIB. Vous le savez, cette dégradation aurait été temporaire exceptionnelle, résultant en grande partie de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, en baisses de cotisations sociales, ce qui représente de l'ordre de 0,9 point de PIB. Après le dépôt du projet de loi de finances, des dispositions fiscales et sociales nouvelles de soutien au pouvoir d'achat ont été annoncées. Constituées principalement de baisses de prélèvements, elles représentent un montant proche de 11 milliards d'euros. Le Gouvernement a alors annoncé des mesures de compensation, qui contiendraient, selon lui, la hausse du déficit à 3,2 points de PIB. Dans ce scénario, la dette publique française augmenterait toutefois, contrairement à ce que prévoit la loi de programmation des finances publiques que vous avez adoptée en décembre 2017. Voilà pour les faits. La Cour constate que la prévision de déficit public du Gouvernement, ainsi contenue à 3,2 points de PIB, est soumise à plusieurs incertitudes. J'en citerai trois. La première tient au fait que le scénario macroéconomique défini en septembre 2018 en loi de finances initiale présente désormais un risque sérieux de ne pas se réaliser. Il table sur une prévision de croissance à 1,7 % pour 2019. Or, depuis le moment où cette prévision a été élaborée, l'environnement macroéconomique s'est dégradé en Europe et dans le monde. Les dernières prévisions de l'INSEE en témoignent ; elles anticipent en effet pour 2018 une croissance de 1,5 %, moins élevée que la prévision initiale de 1,7 %. Deuxième incertitude si une partie des mesures de soutien au pouvoir d'achat annoncées en fin d'année a été votée en loi de finances, la prévision de déficit du Gouvernement n'intègre pas l'impact des dispositions figurant dans la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales, estimé à 3,7 milliards d'euros. Le Gouvernement s'est engagé à le compenser en intégralité ultérieurement ; cela reste à documenter et à concrétiser. Enfin, pour que la hausse du déficit ne dépasse pas la cible de 3,2 points de PIB, les objectifs de dépense des administrations publiques votés dans les lois de finances pour 2019 devront être parfaitement tenus, dans un contexte de ralentissement économique. Que retenir au-delà de ces chiffres ? Les efforts de redressement engagés par la France ces dernières années semblent s'essouffler. S'agissant de la situation de ses comptes publics, l'écart se creuse entre notre

de nos finances publiques par le passé, les pouvoirs publics disposent aujourd'hui de moins de marges de manoeuvre pour soutenir l'activité du pays et protéger nos concitoyens les plus fragiles. À court terme, la Cour estime donc indispensable que le Gouvernement vous présente, dès que possible, des projets de lois financières rectificatives pour l'État et la sécurité sociale. intégrer, de manière sincère et exhaustive, l'ensemble des mesures annoncées par l'exécutif en décembre et les conséquences de l'évolution défavorable de la situation macroéconomique que nous observons depuis l'automne. le Gouvernement devra aussi actualiser la trajectoire des finances publiques figurant dans la loi de programmation pour 2018 à 2022, promulguée en janvier 2018. Certaines de ses dispositions ont en effet été rendues caduques par les décisions budgétaires prises en fin d'année 2018 et l'évolution de la conjoncture. À plus long terme, pour retrouver des marges de manoeuvre budgétaires, pour faire baisser les prélèvements obligatoires et pour réduire sa dette publique, notre pays doit accélérer sa transformation. C'est mon deuxième message. Malgré les constats que je viens de formuler, le propos des juridictions financières aujourd'hui ne se veut pas résigné ; il est au contraire volontairement optimiste. Au travers de nos contrôles, nous avons la conviction que la situation dans laquelle se trouve notre pays n'a rien d'inéluctable. J'en veux pour preuve que certains de nos voisins- j'ai cité à titre d'exemple le cas de l'Allemagne -parviennent, eux, à redresser en profondeur leurs comptes publics. Nous savons aussi, et c'est le coeur de nos travaux, que des marges importantes existent en repensant l'utilité de chaque euro dépensé. Or, selon nous, ces marges sont insuffisamment exploitées. Le rapport public annuel présente justement un certain nombre d'exemples à l'appui de cette observation. Côté dépenses, le rapport explore différentes pistes. S'agissant des pistes de réduction des dépenses, il identifie des possibilités importantes résultant de l'amélioration de la gestion des charges de personnel dans les collectivités publiques. En 2016, la masse salariale par habitant de la commune de Bobigny était, par exemple, supérieure de 34 % à celle des villes de taille comparable. De manière générale, la gestion des ressources humaines de cette collectivité est marquée par des irrégularités, signalées à plusieurs reprises par la chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Autre exemple cité dans le rapport : dans douze communes défavorisées d'Île-de-France, la durée annuelle légale du temps de travail n'est que rarement respectée, exposant les collectivités concernées à des charges non justifiées qui grèvent les budgets communaux, même si, bien évidemment, pour répondre aux aux besoins spécifiques des populations de ces communes défavorisées, il peut y avoir d'autres moyens à mettre en oeuvre. Mieux dépenser aujourd'hui permet aussi parfois de réduire les charges de demain. C'est le sens du chapitre consacré à la politique de prévention des infections associées aux soins, aux soins, appelées maladies nosocomiales. Des progrès indéniables ont été progressivement réalisés pour limiter les contagions, mais, à l'hôpital, un patient sur vingt est encore infecté chaque année. Cette

Il revient aussi aux décideurs d'orienter le mieux possible les moyens publics pour maximiser leur efficacité. La politique des lanceurs spatiaux en est une illustration. Cette politique revêt un caractère stratégique pour la France et pour l'Europe. Elle s'appuie sur le lanceur Ariane 6, développé dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, sur l'initiative de la France. Aujourd'hui, toutefois, ce lanceur ne constitue pas une réponse suffisante aux défis de la concurrence américaine. La Cour recommande donc, d'une part, que les pouvoirs publics français mobilisent davantage leurs partenaires européens pour rendre Ariane 6 plus compétitive et, d'autre part, que cette mobilisation serve à financer prioritairement l'innovation technologique au profit des lanceurs, et non leur fonctionnement courant. Dans ce rapport, la Cour met aussi en évidence que, dans certains domaines, les dépenses n'ont pas toutes vocation à relever du seul secteur public. C'est l'un des messages que porte notre chapitre consacré au contrôle de la sécurité sanitaire de l'alimentation. La Cour y recommande notamment une plus grande participation des professionnels du secteur au financement des contrôles effectués par l'administration. En effet, alors que, en France, leur contribution représente environ 10 % des sources de financement de cette politique, au Danemark, cette proportion atteint près de 47 %. Lorsque les acteurs de la dépense sont multiples, il revient aussi aux pouvoirs publics de les fédérer autour d'un modèle économique clair et solide. C'est la recommandation que nous portons s'agissant de la filière thermale développée dans la région Occitanie. Dans certains cas, ce sont les conditions d'exécution des dépenses publiques qui conduisent à en interroger le principe même. C'est l'interrogation que formule la Cour à l'égard du Mobilier national des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie. Dans le chapitre qui leur est consacré, la Cour met également en évidence des défaillances de gestion inacceptables au sein de ces structures. On peut parfois s'étonner que cela n'émeuve pas, tout particulièrement les responsables de ce service. L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, fait l'objet de critiques du même ordre, elle qui a accumulé, entre 2013 et 2017, près de 508 millions d'euros de pertes d'exploitation. Les pouvoirs publics gagneraient, dans cette situation, soit à accompagner une réorganisation de grande ampleur de l'Agence, soit à envisager la reprise de ses activités par d'autres entités. Côté recettes, la Cour identifie également des marges de progrès. L'une d'entre elles concerne la lutte contre toutes les formes de fraudes sociales et fiscales. La fraude au travail détaché fait, par exemple, l'objet d'un chapitre spécifique. Celui-ci révèle que, si l'arsenal juridique français est aujourd'hui suffisant, notre pays a tardé à le mettre en place pour faire face aux différents types de fraudes, parfois très sophistiqués. Nous recommandons également qu'une meilleure utilisation soit faite des outils existants, tant sur le volet des contrôles- ils peuvent encore être améliorés -que sur celui des sanctions. Enfin, faire le meilleur usage des fonds dont bénéficient les projets publics, c'est le sens des recommandations formulées à l'encontre de la gestion des fonds européens structurels et d'investissement en outre-mer. La Cour chiffre à 4,8 milliards d'euros le montant reçu de l'Union européenne par la France, entre 2014 et 2020, soit une somme très élevée. En contrôlant les plus gros projets financés, elle a constaté de belles réussites, qu'elle mentionne, mais elle déplore aussi des difficultés de gestion ayant conduit au gaspillage d'une partie de cette ressource. Voilà pour quelques exemples et pistes de réflexion ouvertes par ce rapport.

une recette miracle, susceptible de dégager des milliards d'euros d'économies. Mais les petits ruisseaux forment les grandes rivières ... Pour parvenir à ces grandes rivières, il faut aussi que le courant soit bien canalisé, c'est-à-dire que les réformes soient correctement et durablement engagées. C'est le troisième et dernier message que je souhaite formuler devant vous. Nous en sommes les témoins privilégiés lors de nos contrôles, nombre d'organismes publics engagent des processus courageux de transformation. Toutefois, la Cour constate trop souvent leur caractère incomplet. Pour que ces démarches portent pleinement leurs fruits, il faut en effet s'attaquer aux causes des déséquilibres financiers ou des inefficiences de la dépense. Notre rapport public offre notamment trois exemples à l'appui de ce message. Le premier porte sur le réseau des trains Intercités. Pour enrayer le déclin de ce réseau, l'État a engagé une réforme profonde qui conduira, d'ici à 2020, au transfert de dix-huit lignes aux régions. La Cour note que cette réforme n'a pas traité tous les enjeux auxquels est confronté le réseau : des incertitudes demeurent quant à l'avenir de son modèle économique, atypique au plan européen, en particulier face à l'ouverture à la concurrence du secteur qui interviendra à partir de 2023. Très hétérogène, le réseau offre, en outre, une qualité de service inégale. Enfin, les modalités de gouvernance entre l'État, l'exploitant et les régions demeurent, elles aussi, fragiles. qui a fait l'objet de nombreux contrôles de la Cour des comptes, constitue un autre exemple développé dans ce rapport. Notre juridiction y souligne les progrès accomplis par l'entreprise, dont témoignent ses bons résultats d'audience. la transformation engagée n'est pas allée suffisamment loin pour assainir pleinement la situation de l'entreprise et lui permettre d'affronter les mutations majeures de son activité. Des évolutions de structure restent à opérer, notamment pour réduire ses charges de personnel ou pour moderniser ses relations sociales. Alors que le chantier de réhabilitation de la Maison de la radio entre dans sa treizième année, la situation financière de Radio France demeure fragile. Accompagner la transformation publique en remettant à plat l'activité des services : c'est l'enjeu, enfin, du chapitre dédié aux urgences hospitalières, qui réitère des messages récurrents de la Cour des comptes. Alors que la demande ne cesse de croître, notre institution constate que de 10 % à 20 % des recours aux urgences auraient pu être traités en médecine générale. En bout de chaîne, les services des urgences apparaissent ainsi comme le réceptacle des dysfonctionnements de l'articulation du milieu hospitalier avec la médecine de ville. Bien sûr, les différents exemples cités tendent à donner le sentiment que les actes tardent à venir, quand bien même les causes des difficultés sont depuis longtemps identifiées. Pourtant, notre rapport public annuel est aussi l'occasion d'adresser des « coups de chapeau » à des transformations réussies. Nous le faisons cette année à propos de deux sujets, celui de la réforme des avoirs bancaires et des contrats d'assurance vie en déshérence et celui du service militaire adapté en outre-mer. Le suivi annuel de nos recommandations est aussi pour nous une source de satisfaction ; j'aimerais m'y arrêter un bref instant. Le suivi statistique que nous réalisons chaque année montre que 72 % des recommandations formulées entre 2015 et 2017 par la Cour des comptes ont été totalement ou partiellement mises en oeuvre par les administrations. Cette proportion est encore supérieure pour les chambres régionales et territoriales des comptes, où elle s'élève à 79 %. Ces chiffres incluent le pourcentage de recommandations totalement mises en oeuvre, qui atteint 24 comptes et 4 % pour les chambres régionales. Vous trouverez à la fin du deuxième tome de notre rapport public annuel de nombreuses illustrations de ce suivi. Nous y constatons par exemple, au titre des recommandations que nous avons formulées par le passé, les progrès réalisés pour renforcer la lutte contre la fraude dans les transports urbains en Île-de-France. Nous nous réjouissons aussi du recentrage du dispositif des contrats aidés. Nous saluons, enfin, le transfert aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les Urssaf, de tâches que le régime social des indépendants n'arrivait plus à assumer. Je pourrais multiplier les exemples, mais je vous renvoie à la lecture du tome II de notre rapport. Toutes les recommandations qui figurent dans cette édition 2019 feront l'objet du même suivi : nous retournerons donc, dans quelques années, constater, dans les organismes et les administrations qui ont été cités ce matin, les progrès qu'ils auront réalisés ou non. Monsieur monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, malgré les progrès accomplis, en ce début d'année, la situation des finances publiques de notre pays demeure fragile, marquée par de fortes incertitudes. Les rapports que nous publions année après année peuvent donner le sentiment que rien ne change. Ce n'est pas notre message ni notre conviction. Au fil des contrôles que nous effectuons, il nous appartient évidemment de souligner ce qui ne fonctionne pas de formuler des recommandations utiles pour remédier aux dérives de gestion que nous constatons, mais notre activité nous conduit aussi à relever des progrès, à identifier des voies nombreuses de transformation et à observer le professionnalisme, l'engagement et le sens du service des agents qui concourent à la modernisation de l'action publique. Notre mission d'information et d'explication, nous l'accomplirons cette année encore dans un contexte de plus en plus exigeant, à une époque où la parole publique, quel qu'en soit l'auteur, est mise en doute et où la production d'une information objective est menacée par la propagation de fausses nouvelles. Cette exigence nous invite à un effort permanent de transparence, d'explication, d'écoute, donc d'adaptation de nos pratiques. Comme celles qui l'ont précédée, l'année 2019 offre aux juridictions financières de nouveaux chantiers de nouveaux chantiers de transformation. Ils visent, pour beaucoup d'entre eux, à favoriser l'appropriation de nos travaux par leurs différents destinataires, en particulier par le Parlement. J'ai mentionné à ce titre la modification de notre calendrier de publication. Nous ambitionnons aussi d'améliorer notre politique de publication, en continuant d'offrir aux citoyens des supports de communication plus diversifiés, plus pédagogiques, plus innovants. Le rapport public annuel qui sera publié l'année prochaine devrait par exemple évoluer par rapport à la version que nous vous remettons aujourd'hui. Il devrait nous permettre de traiter notamment un thème dominant, en l'espèce celui du numérique au service de la transformation de l'action publique. Je l'ai dit, notre but, au travers de ces évolutions, est de vous être toujours plus utiles, afin que nous contribuions ensemble, chacun dans nos missions, dans notre positionnement institutionnel, à la transformation du service public pour rendre l'action publique

comme chaque année, M. le Premier président de la Cour des comptes présente au Parlement le rapport public annuel de celle-ci. C'est un moment solennel pour notre assemblée, qui symbolise, davantage qu'il ne résume, la richesse de nos relations avec la Cour En effet, il est désormais loin le temps où le rapport public annuel constituait l'unique synthèse des travaux de la Cour des comptes dont les parlementaires pouvaient s'inspirer pour réformer l'action publique. Comme le lui prescrit notre Constitution, la Cour des comptes assiste tout au long de l'année le Parlement, ainsi que le Gouvernement, dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que, de façon plus générale, dans l'évaluation des politiques publiques.

commande régulièrement à la Cour des comptes des enquêtes susceptibles d'éclairer l'ensemble des sénateurs sur des sujets d'intérêt général. C'est une contribution utile à l'information des citoyens.

Nous les entendrons de nouveau dans quelques jours sur l'important sujet de la dette des entités publiques ou encore, au début du mois de mars, sur la Caisse de garantie du logement locatif social. Leur expertise alimente les travaux et réflexions de nos rapporteurs spéciaux, tout comme la Cour des comptes s'inspire aussi des nombreuses informations et pistes de travail contenues dans les rapports du Sénat. À cet égard, je voudrais souligner ce qui, dans ce rapport annuel, attire plus particulièrement l'attention de la commission des finances. En premier lieu, il s'agit bien évidemment du chapitre relatif à la situation d'ensemble de nos finances publiques, qui confirme ce que nous ne savons que trop, à savoir que la loi de finances pour 2019 ne prend que très partiellement en compte l'incidence budgétaire des mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages adoptées, dans les conditions adoptées, dans les conditions que l'on sait, en fin d'année. Pour être précis, leur coût est de l'ordre de 11 milliards d'euros tout de même, mais seulement 4,1 milliards d'euros de mesures de compensation ont été annoncées, sans avoir encore été prises Il s'agit notamment de la restriction de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, de la nouvelle taxe sur les grands acteurs de l'internet, ou encore, soyons clairs, des mesures d'économie sur les dépenses de l'État qui restent à concrétiser. Le Gouvernement passe sous silence les fragilités de nos perspectives macroéconomiques dans un contexte de ralentissement européen et mondial. La Cour des comptes mentionne un scénario des finances publiques « préoccupant » et « estime indispensable que le Gouvernement présente, dès que possible, des projets de lois financières rectificatives, pour l'État et pour la sécurité sociale, intégrant de manière exhaustive et sincère l'ensemble des mesures annoncées ainsi que les conséquences de l'évolution de la situation macroéconomique Dans sa réponse, le Gouvernement temporise en renvoyant au programme de stabilité d'avril, qui sera présenté à la Commission européenne mais qui ne remplace pas un texte budgétaire soumis au Parlement L'existence d'un grand débat fiscal ne saurait masquer la responsabilité du Gouvernement de revenir devant les parlementaires le plus rapidement possible pour préciser le cadrage de nos finances publiques, et ce avant toute présentation de la trajectoire de nos finances publiques devant la Commission européenne.

de la majorité de nos partenaires européens, et que la dette publique rapportée au produit intérieur brut devrait encore augmenter en 2019. Le niveau relativement élevé de la croissance- 1,5 % à 1,7 % en 2018, selon les estimations -n'a pas été mis à profit pour commencer à réduire le poids de la dette publique. Lors de son arrivée en juin 2017, le nouveau gouvernement avait demandé à la Cour des comptes un « audit » des finances publiques, dans lequel celle-ci s'alarmait du fait que « sans mesures nouvelles de redressement, le déficit public dépasserait de 0,4 point de PIB l'objectif, pour atteindre 3,2 points Aujourd'hui la Cour des comptes note sobrement que « le Gouvernement a annoncé vouloir adopter courant 2019 des mesures de hausse de prélèvements obligatoires et de baisse des dépenses de l'État [ ...] afin de maintenir à 3,2 points de PIB le déficit prévu L'objectif semble être non plus de réduire le déficit en dessous de 3 % du PIB, mais de ne pas l'augmenter davantage ! Monsieur le Premier président, la Cour frôle la complaisance ; c'est inhabituel J'en viens maintenant à d'autres assertions du rapport public annuel qui font écho aux observations formulées par nos rapporteurs spéciaux sénatoriaux. Elles figurent principalement dans le suivi des recommandations, deux chapitres seulement constatant des progrès, six insistant sur les réformes à poursuivre et deux alertant. Parmi les points positifs, la Cour des comptes dresse le bilan de l'application de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Concernant ces derniers, le rapport fait état du maintien d'un stock de contrats en déshérence à un niveau élevé, en dépit des efforts réalisés par les assureurs. Je tiens à souligner que notre assemblée s'est saisie de ces sujets depuis de nombreuses années : notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, avait ainsi pointé le problème des contrats de retraite complémentaire, tenant en particulier au fait qu'ils ne prévoient pas d'échéance, en introduisant dans la loi dite « Sapin II » une disposition à ce sujet. De nouveaux amendements ont également été adoptés sur l'initiative de plusieurs sénateurs à l'occasion de l'examen du projet de loi PACTE pour inciter davantage les assureurs à rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance vie. Autre motif de satisfaction, la Cour des comptes constate les bons résultats du service militaire adapté en matière d'insertion socioprofessionnelle des jeunes dans tous les territoires d'outre-mer, et ce en dépit de l'augmentation importante des effectifs qu'il a connue depuis 2010. Elle relève toutefois la nécessité d'améliorer le taux d'encadrement, d'axer davantage ce dispositif sur les formations longues et d'en renforcer la gouvernance. Nos collègues Nuihau Laurey et Georges Patient ne manqueront pas d'être attentifs à ces conclusions, puisqu'ils rendront compte dans quelques jours devant la commission des finances de leur contrôle sur le service militaire adapté, qui les a amenés à Mayotte. Parmi les sujets sur lesquels la Cour des comptes insiste figure le contrôle de la sécurité sanitaire de l'alimentation -sujet sensible et d'actualité s'il en est -, dont la Cour des comptes estime que les progrès sont à consolider, faisant notamment référence à l'excellent rapport d'Alain Houpert et de Yannick Botrel sur ce sujet.

avant puis au moment de l'affaire dite « Lactalis », et nous poursuivrons, avec l'appui des analyses de la Cour des comptes, cet engagement vigilant quant aux moyens donnés à la protection de la santé des consommateurs. Dans le suivi des recommandations, la Cour des comptes souligne que le chantier de réhabilitation de la Maison de la radio a connu de nouveaux retards et que ses coûts ont encore augmenté. Elle pointe les risques et les incertitudes persistantes concernant ce chantier et recommande une clarification des conditions de financement de la fin des travaux. Dans son rapport spécial pour 2019, notre collègue Roger Karoutchi avait concentré ses observations sur ces mêmes risques et incertitudes. Ces conclusions rejoignent donc largement celles de notre rapporteur spécial. Enfin, nous ne manquerons pas d'utiliser les travaux que nous livre la Cour des comptes en vue de nos prochaines auditions de responsables publics. Tout comme le rapport sur la Banque de France avait fourni l'occasion d'interroger le gouverneur sur les missions confiées à l'institution qu'il dirige, nul doute que les recommandations de la Cour des comptes concernant la nécessité pour l'Agence française de développement, l'AFD, de concilier l'extension de son champ d'intervention avec une amélioration de son pilotage financier alimenteront la réflexion de nos collègues rapporteurs spéciaux Yvon Collin et Jean-Claude Requier et les débats devant notre commission à l'occasion de l'audition prochaine du directeur général de l'AFD. En conclusion, je ne peux que souhaiter, monsieur le Premier président, que nos relations de travail avec la Cour des comptes se poursuivent selon les modalités qui ont été définies ces dernières années, la Cour aidant le Parlement à contrôler l'action du Gouvernement et répondant aux demandes d'enquêtes formulées par les sénateurs, ceux-ci, dans leurs fonctions législatives et de contrôle, décidant des suites qu'ils entendent y apporter. La

des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, chaque année, les termes de l'article 47, alinéa 2, de la Constitution trouvent une traduction dans la présentation du rapport public annuel de la Cour des comptes, traduction qui est bien loin d'être la seule. Je saisis l'occasion qui m'est ici donnée pour saluer de nouveau, à la suite du président Larcher, la qualité de l'enquête récemment remise à la commission des affaires sociales sur les président, d'une contribution tout à fait remarquable au débat qui s'est ouvert sur la transformation du système de santé, mais surtout d'un appel à une cohérence dans les choix publics qui se fait plus rare encore dans les temps que nous connaissons. Je ne doute pas que les enquêtes à venir, qui porteront sur l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, et sur la politique en matière de lutte contre le VIH-sida seront tout aussi passionnantes. Dans le rapport public annuel qui nous est aujourd'hui présenté, la Cour des comptes évoque de nombreux sujets sociaux, qu'il s'agisse du travail détaché, des infections associées aux soins, de l'action sociale de l'Agirc-Arrco, voire du thermalisme ... J'y vois la marque d'un intérêt justifié, notamment, par leur enjeu pour les finances publiques. S'agissant de la situation d'ensemble des finances publiques, la Cour des comptes évoque des « prévisions particulièrement fragiles la compétitivité et l'emploi, le CICE, la dégradation de la conjoncture internationale et les mesures d'urgence sociale adoptées avant Noël introduisent de fortes incertitudes sur la trajectoire budgétaire. Alors certes, dans ce paysage d'ensemble plutôt inquiétant, les comptes sociaux peuvent sembler un peu plus « brillants » que les autres comptes publics. Néanmoins, là aussi, de fortes incertitudes demeurent. les comptes sociaux sont, plus encore que les autres, sensibles à la conjoncture économique. Ensuite, comme l'a souligné le rapporteur général de la commission des affaires sociales, Jean-Marie Vanlerenberghe, de non-compensation des mesures d'urgence de l'automne, le solde de la sécurité sociale s'établirait, en négatif, à 2,8 milliards d'euros, loin du retour à l'équilibre annoncé en octobre dernier. Une partie au moins des économies envisagées par le Gouvernement en 2020 reste hypothétique. Je pense aux quelque 3 milliards d'euros que devait rapporter une nouvelle année de gel de nombreuses prestations sociales, en particulier les pensions de retraite et les allocations familiales. Après la censure du Conseil constitutionnel, le Gouvernement inscrira-t-il, dans le contexte social actuel, de telles mesures dans le prochain projet Le cas échéant, le Parlement votera-t-il ces dispositions ? Il est difficile, à ce stade, d'avoir des certitudes. Dans ce contexte, la Cour des comptes appelle le Gouvernement à présenter au Parlement des projets de lois financières rectificatives, ainsi qu'à réviser la trajectoire budgétaire de la France dans le cadre d'une nouvelle loi de programmation des finances publiques. La commission des affaires sociales adhère à cette logique. Elle souhaite que ces futurs projets de loi appliquent le principe de compensation : les mesures de l'automne étaient des réponses de l'État à une crise politique et sociale, et non des mesures concernant la sécurité sociale. Elle souhaite également que ces futurs projets de loi révisent d'ores et déjà les coupes programmées de TVA en direction de la sécurité sociale, dont nous avons dénoncé le caractère irréaliste dès l'automne dernier, afin de ne pas compromettre les perspectives d'apurement complet de la dette de la sécurité sociale à l'horizon 2024. Nous avons le devoir de ne pas léguer le « trou de la sécu » à nos enfants. De plus, la CADES, doit disparaître, l'Agence France Trésor, elle, demeure ... Je voudrais ensuite évoquer brièvement les différents sujets abordés par la Cour des comptes relevant de la commission des affaires sociales, sans pouvoir bien sûr rendre totalement justice à leur intérêt.

En raison notamment de coûts de structure trop importants et de la perte de marchés publics, l'agence enregistre des pertes colossales. Selon la Cour des comptes, les subventions exceptionnelles versées chaque année à l'AFPA posent, outre la question de leur conformité au droit de la concurrence, celle de la bonne gestion d'une structure qui a jusqu'à présent échoué à se réformer de manière efficace. Sous l'égide d'une nouvelle équipe de direction, l'AFPA a lancé un plan de transformation qui apparaît comme un plan de la dernière chance, ainsi que l'avait souligné notre collègue Michel Forissier dans son rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2019. Comme le souligne la Cour des comptes, la réussite de ce plan sera tributaire d'un recentrage de l'AFPA sur son coeur de métier et de la fixation par l'État d'objectifs clairs conditionnant l'octroi de toute nouvelle aide. La Cour des comptes s'attarde également sur la lutte contre la fraude au travail détaché, dont la commission des affaires sociales a eu à traiter à l'occasion de chaque texte visant à la renforcer, c'est-à-dire presque chaque année depuis 2014. Si l'arsenal juridique s'est ainsi renforcé, la Cour des comptes souligne que les sanctions administratives et pénales créées par le législateur ne sont pas suffisamment appliquées. Enfin, il est impératif de renforcer la coopération européenne en la matière. On notera toutefois avec intérêt que, si la France figure parmi les pays qui reçoivent le moins de demandes, ses délais de réponse sont parmi les plus longs. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, la Cour des comptes recommande au ministère du travail d'accélérer les délais de réponse aux demandes d'informations émanant de nos partenaires européens. Le modèle économique de l'Établissement français du sang Le modèle économique de l'Établissement français du sang se trouve aujourd'hui fragilisé par les mutations profondes de la filière du sang, à l'heure où la concurrence s'intensifie dans le secteur des médicaments dérivés du sang. Le marché mondial du plasma, en pleine expansion et régulièrement en situation de pénurie, est désormais dominé à 85 % par les dons américains, rémunérés, qui n'offrent pas les mêmes garanties éthiques et de sécurité. Vous appelez à conforter notre modèle de don, gratuit, bénévole et anonyme, non seulement en réduisant les coûts de la collecte du plasma, mais également en indemnisant mieux et de façon éthique le don du sang en France. Il est temps, à mon sens, que nous évoluions sur cette question, afin de ne plus nous retrouver contraints d'importer des produits américains dont les conditions de collecte s'éloignent de nos standards éthiques. de lutte contre les infections associées aux soins, le chapitre dresse un constat préoccupant sur la menace de l'antibiorésistance en France.

Notre arsenal thérapeutique contre les infections nosocomiales s'en trouve lourdement fragilisé. Or 93 % de la consommation d'antibiotiques résulte de prescriptions faites en ville. Ne nous leurrons pas, des médecins continuent de prescrire des antibiotiques pour le traitement d'infections virales des voies aériennes, notamment pendant les épisodes grippaux Comme le proposent nos collègues Yves Daudigny et Michel Amiel, qui ont interpellé le Gouvernement sur ce sujet, oeuvrons résolument pour la juste prescription.

d'écarter la piste d'une infection bactérienne et de convaincre les patients, résultat à l'appui, de l'inutilité d'une antibiothérapie.

Toujours plus sollicités, soumis dans certains établissements à des tensions devenues insupportables, les services des urgences accueillent une large part de soins non programmés qui pourraient tout aussi bien- et probablement même mieux -être pris en charge en ville. Il importe de recentrer chacun des acteurs du système de soins sur le coeur de sa compétence, ce qui permettra de renforcer la qualité des soins comme la satisfaction des professionnels. Force est cependant de constater que, si ces éléments sont largement connus et documentés, la situation n'évolue pas. pas. L'actualité récente nous a fourni plusieurs exemples tragiques des difficultés rencontrées par les établissements les plus exposés. C'est que, comme bien souvent, les constats sont mieux partagés que les remèdes. Je mets en garde contre toutes les solutions de « bricolage » qui viendraient réformer les urgences sans vision d'ensemble, à l'image du forfait de réorientation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. C'est aujourd'hui à une refondation globale des urgences que nous devons nous atteler, et plus généralement à une réflexion approfondie sur le partage des tâches entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, assorti, bien entendu, des moyens adaptés de part et d'autre.

pleinement dans les préoccupations du Parlement, les éclairent et les complètent, pour un meilleur contrôle de l'action du Gouvernement. Monsieur le

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,

» de la normalisation comprend un numéro 10, l'AFNOR, qui est la plaque tournante, et de bureaux de normalisation sectoriels agréés. Chacun doit tenir son rôle. Le présent amendement vise à rendre plus lisible la composition de cette équipe de France et à faciliter des coopérations avec les organisations européennes ou internationales de normalisation.

d'éviter que l'on alourdisse inutilement les coûts de traduction à la charge de l'AFNOR en lui imposant la traduction systématique de toutes les normes qu'elle publie, y compris celles qui ne seront pas utilisées en version française, du fait des pratiques d'une filière industrielle ou de services très internationalisés. Dans ce dernier cas, on lui permettrait de n'en traduire qu'un résumé, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

les coûts de production, assorti d'un engagement social et environnemental et d'une obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d'une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique. Aujourd'hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables »- lait équitable, fruits équitables, etc. -, mais ils recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements pas toujours conformes aux principes du commerce équitable énoncés à l'article 94 de la loi du

Comme pour les produits dits « bio », qui doivent respecter la réglementation sur l'agriculture « biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrite à l'article 94 de la loi ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

l'avis du Gouvernement ? Le règlement relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires contient des dispositions qui permettent aux professionnels d'utiliser des informations facultatives sur les denrées alimentaires, dans la mesure où ces informations sont vraies et loyales- c'est l'article 36 de ce règlement. des dispositions générales du code de la consommation prohibent les pratiques commerciales déloyales : les articles L. 121-1 et suivants sanctionnent les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros,

M. Jean-Louis Tourenne. Après un premier amendement prévoyant une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées, rejeté par la majorité sénatoriale, le groupe socialiste et républicain va présenter une série d'amendements qui forment un dispositif global de développement de la démocratie et de la justice sociale dans l'entreprise. Notre groupe a considéré, en effet, que l'objectif pompeusement affiché par le Gouvernement de « mieux partager la valeur » n'était pas au rendez-vous de ce projet de loi- j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier soir. Fonder ce meilleur partage de la valeur sur la seule épargne salariale omet les sujets centraux que sont le partage entre dividendes et salaires, les écarts de salaires et la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise. La réduction des écarts de richesse et la lutte contre les inégalités participent de la cohésion nationale, comme sont venus nous le rappeler le mouvement dit des « gilets jaunes » et sa revendication principale de justice sociale. Celle-ci passe, notamment, par la réduction des écarts de salaires, dont l'ampleur n'est plus admissible admissible ni socialement admise. Dans cette perspective, nous proposons de renforcer la démocratie dans les grandes entreprises en matière de contrôle des rémunérations. Celui-ci doit être double : par les actionnaires

à travers leurs institutions représentatives. Cet amendement vise en effet à instaurer un avis conforme du comité social et économique préalable, avant l'approbation de la résolution annuelle sur les rémunérations par l'assemblée générale des actionnaires.

monsieur Bourquin, vous invoquez la transparence pour les hauts salaires dans les entreprises, mais où est la transparence

visent à protéger les entreprises des dérives de la financiarisation de l'économie en faisant primer l'emploi et le long terme sur le cours de la bourse. L'amendement n° 334 rectifié tend à interdire aux entreprises de s'endetter pour verser des dividendes aux actionnaires, pratique malheureusement trop courante. Ainsi, GRDF a versé, en 2017, 1 milliard d'euros de dividendes, pour un résultat de 150 millions

Selon le rapport qu'Oxfam a consacré aux entreprises du CAC 40, « si l'on ramène le montant des dividendes versés au montant des bénéfices réalisés, la France est alors la championne mondiale entre 2005 et 2015, ce sont les entreprises du CAC 40 qui ont reversé la plus grande part de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes ». Ces entreprises françaises sont ainsi et « de loin les plus gros payeurs de dividendes en Europe continentale » ; les dividendes qu'elles versent sont chers collègues, nous vous proposons donc de rééquilibrer le rapport entre dividendes et salaires, pour plus de justice sociale et dans l'intérêt même de la pérennité des entreprises. J'ajoute que c'est l'investissement

dont nous avons parlé hier dans cet hémicycle, elle a versé, en 2016, « quinze fois plus de dividendes à ses actionnaires que ce que l'entreprise a fait de bénéfices ». La priorité donnée à la distribution de dividendes est également au détriment de l'investissement, favorisant une logique de court terme. Entre 2012 et 2014, les entreprises du CAC 40 ont ainsi augmenté les dividendes de 44 %, tout en diminuant leur capacité d'investissement

Louise Michel : « Les élites n'ont pas conscience de ce qui se passe. [ ...] Après la crise de 2008, il y a eu une conscience [ ...] de ce qu'il fallait faire : réglementer certains secteurs financiers [ ...]. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La réglementation financière recule ici ou là [ ...]. Le laxisme revient. »

Mais la nature a horreur du vide, et la liberté trouve toujours son chemin ... Vous vous définissez comme un libéral : le plus grand libéral que je connaisse en France, c'est le consommateur qui pousse son caddie au supermarché.

Bien que son principal objet soit de pérenniser une société, le fonds de pérennité appartient à la grande famille des fondations et des fonds. Il n'est donc pas approprié de codifier les articles qui s'y rapportent dans le code de commerce.

Le caractère hybride du fonds de pérennité est au coeur du projet : c'est dans la réalisation de cette double mission que réside toute la valeur ajoutée de cette structure. C'est pourquoi la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoyait d'autoriser le fonds de pérennité à réaliser ou à financer des oeuvres ou des missions d'intérêt général.

qui ont une finalité philanthropique. Elle aura en premier lieu une vocation économique et de garantir la stabilité des entreprises sur le long terme. » Je souscris totalement

le groupe Bolloré soutient la recherche médicale l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Il y a également du mécénat indirect, avec des sociétés qui créent des fondations distinctes : c'est ainsi que la fondation Michelin contribue à hauteur de 13 millions d'euros au financement de projets et que la fondation Monoprix soutient une association d'aide aux femmes sans domicile fixe.

Il semble que de nombreux entrepreneurs souhaitent non seulement transmettre les titres de leur entreprise à une structure qui pérennise les valeurs morales et économiques qu'ils ont développées, mais également financer des missions philanthropiques de manière directe, grâce aux bénéfices produits. La valeur ajoutée du fonds de pérennité réside précisément dans la poursuite de cette double mission. Cette structure, qui s'inspire des meilleurs exemples européens, notamment de l'exemple danois, permet d'inscrire de manière efficace le développement économique d'une entreprise au coeur de son environnement social et environnemental. Supprimer cette dimension contraindrait inutilement les entrepreneurs intéressés à créer deux structures entièrement séparées et les empêcherait d'utiliser directement les fruits de leur société pour le développement d'activités nouvelles. Je mets aux voix l'amendement

À l'issue des opérations de liquidation, l'actif subsistant, lequel peut comprendre les titres initialement apportés, sera transféré soit à un bénéficiaire désigné par les statuts, soit à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation. La difficulté naît du cas de dévolution de l'actif à une personne qui n'est pas un organisme d'intérêt général. En l'état actuel des textes, il semble que la possibilité de transférer l'actif net à un bénéficiaire désigné dans les statuts, par exemple un descendant du fondateur, non seulement soit en contradiction avec l'idée d'affectation irrévocable des titres, mais en outre permette que les titres fassent l'objet, à plus ou moins brève échéance, d'une transmission à titre gratuit à une personne physique.

de l'argument selon lequel l'application des droits de mutation à titre gratuit serait dissuasive, il semble que cette seconde donation, selon la rédaction des statuts, puisse correspondre à la qualification de dotation graduelle, ou résiduelle, ce qui autoriserait la déduction des droits acquittés lors de la première donation. Par

sous-amendement. Dès lors que le bénéficiaire est désigné par les statuts, je ne vois pas quel problème poserait le transfert de l'actif net du fonds. Imaginons qu'une entreprise de taille intermédiaire familiale tente l'aventure du fonds de pérennité, avant de se rendre compte que ce nouveau cadre est trop rigide et ne lui permet pas de s'adapter aux aléas économiques et de pérenniser des emplois. Il me semble que les statuts pourraient prévoir, pour ce cas de figure, une dissolution du fonds. En pareil cas, quoi de plus normal que de transférer l'actif à un membre de la famille qui a créé l'entreprise et ses éventuelles filiales ?

Cet amendement vise à répondre aux questions que M. le sénateur Bargeton vient de soulever. Nous proposons de confirmer que l'éventuelle transmission de l'actif net du fonds de pérennité à la suite de la liquidation de celui-ci est, comme toute libéralité consentie par une personne morale, assujettie aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun.

Il s'agit d'étendre aux représentants des salariés actionnaires l'exception prévue pour les représentants des salariés en matière de règles de parité.

Certes, cela va dans le sens d'une plus forte représentation des salariés dans les conseils d'administration, mais il faut selon nous aller plus loin. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'assurer une présence minimale de deux administrateurs salariés dans tous les conseils d'administration, à l'exception, bien sûr, de ceux qui n'en comprennent que trois.

À l'instar de nombre des dispositions de ce projet de loi, cet article est symptomatique de la politique du Gouvernement, qui présente comme des réformes majeures ce qui constitue en réalité des avancées médiocres.

À l'évidence, elle ne permettra pas d'infléchir la gouvernance d'entreprise vers une prise en compte accrue du long terme. Nous proposons donc, sur la base des comparaisons européennes, de fixer un principe clair et ambitieux, sans s'en tenir à une valeur absolue ne tenant pas compte des proportions au sein du conseil d'administration : un tiers d'administrateurs salariés d'administration, quel que soit le nombre d'administrateurs non salariés. Les administrateurs salariés sont la voix de l'intérieur : ils connaissent certaines réalités industrielles, économiques et sociales de l'entreprise que les autres administrateurs n'ont pas toujours à l'esprit au moment de prendre des décisions qui engagent l'avenir de celle-ci. Ils sont les gardiens d'une bonne gouvernance, soucieuse du long terme, dépassant l'horizon de la seule performance financière de court terme. Il est donc essentiel, à l'heure où les entreprises sont de plus en plus enfermées dans la spirale du court-termisme que des enjeux comme la question environnementale sont cruciaux, d'augmenter de façon nette le nombre d'administrateurs salariés dans les conseils, à l'instar de ce qui se pratique en Allemagne et dans la plupart